La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 17 février 2022 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ?

Monsieur le président, monsieur le rapporteur- je suis heureux de

les sénateurs, nous examinons aujourd'hui le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette ordonnance a pour principal objectif d'attirer davantage de personnes dans la fonction publique communale, au service des communes et des administrés de Polynésie. Nous savons combien, en Polynésie française, archipel du Pacifique aussi étendu que l'Europe- on le rappelle souvent -, riche de ses 48 communes des îles du Vent, des îles Sous-le-Vent, des îles Marquises, des îles

exceptionnelles. Ici encore, je veux remercier les maires pour leur action au quotidien, ainsi que les agents du service public qui sont à leurs côtés. Revenons un instant sur la genèse de cette ordonnance dédiée à la fonction publique des communes polynésiennes. À la suite d'un mouvement de grève des fonctionnaires communaux en 2017, des négociations se sont tenues entre l'État, les élus communaux et les organisations professionnelles. Ayant abouti à plusieurs propositions,

Après avis du Conseil d'État, l'ordonnance a été adoptée en conseil des ministres le 8 décembre dernier. Tout au long de ce processus, notre souci a été de moderniser et de rendre plus attractive la fonction publique communale, et ainsi de répondre aux attentes manifestées lors du mouvement social de 2017. La position du Gouvernement a été de faire bénéficier les fonctionnaires des communes de Polynésie française des avancées introduites par les différentes lois relatives à la fonction publique depuis 2011, tout en tenant compte et en intégrant des spécificités locales. locales. Que contient l'ordonnance ? Elle offre avant tout un cadre législatif et réglementaire clair, adapté et sécurisant. Les garanties accordées aux fonctionnaires sont renforcées. Ainsi, la liste des motifs ne pouvant donner lieu à discrimination est complétée par l'ajout de l'identité de genre, la situation de famille et l'état de grossesse. Le principe d'interdiction des agissements sexistes et du harcèlement sexuel est également repris. Les mesures discriminatoires à l'égard des fonctionnaires qui relatent ou témoignent de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou de conflits d'intérêts sont interdites. Le fonctionnaire a désormais droit au temps partiel thérapeutique, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours, au congé de solidarité familiale et au congé pour activité dans la réserve. À l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est réintégré lorsqu'aucun emploi n'est vacant. La protection fonctionnelle dont les agents publics peuvent bénéficier pour eux et leurs proches est enfin renforcée. Les nouvelles règles concernant le cumul d'activités ou l'exercice d'activités privées après la cessation d'une fonction publique et la création d'un référent déontologue sont étendues en Polynésie française. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est lui aussi renforcé. Sa saisine est désormais obligatoire sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif à la fonction publique des communes de Polynésie Tout au long de la concertation, nombre de propositions formulées au niveau local ont été retenues. J'en citerai quelques-unes : le recrutement d'agents contractuels pour remplacer un fonctionnaire en disponibilité ou en détachement de courte durée- cette demande répond à une particularité locale permettant d'accorder aux agents communaux des disponibilités de quelques jours ou semaines pour participer à des événements culturels ou sportifs l'élection autonome des membres représentant les communes au Conseil supérieur de la fonction publique ; la création d'une commission consultative paritaire pour les agents contractuels ; la suppression des limites d'âge au recrutement ; l'extension du congé parental aux trois ans de l'enfant, contre deux ans ; la réouverture, puis la prorogation du droit d'option pour certains agents contractuels ; la suppression du renvoi à un décret pour l'aménagement horaire pour allaitement, dans la mesure où ce droit est déjà garanti par un arrêté du haut-commissaire. la composition des instances paritaires a été adaptée pour répondre aux difficultés de déplacement liées à l'insularité et l'éloignement géographique. Dans le cadre de l'examen du texte au Sénat, il nous semble important de revenir sur plusieurs dispositions adoptées par la commission des lois. lois. Le Gouvernement a donc déposé plusieurs amendements. Ils visent tous à protéger, accompagner et saluer l'engagement des fonctionnaires des communes de Polynésie française. J'aurai l'occasion de les présenter lors de la discussion des articles. Notons néanmoins que le Gouvernement n'a pas déposé d'amendement sur tous les points

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes

de caducité. Il ne serait pas acceptable que le Parlement attende jusque-là pour débattre de sa ratification. La réforme du statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française, portée par l'ordonnance, était en effet attendue

s'est alors ouverte une longue période de concertation entre le Gouvernement et les instances locales- manifestement, elle n'a pas été suffisamment longue, puisque le Gouvernement demande

le statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française au regard, à la fois, des évolutions législatives intervenues dans le droit de la fonction publique territoriale depuis 2011 et des revendications exprimées en mai 2017. La commission a constaté des avancées pour les fonctionnaires communaux communaux de Polynésie française, dont certains droits sont désormais alignés sur le statut de la fonction publique territoriale. Citons, à titre d'exemple, le temps partiel thérapeutique ou encore le congé de paternité. La commission a également salué l'assouplissement des modalités de représentation des élus locaux au sein des instances paritaires. Enfin, des mesures telles que le remplacement de la notation par une appréciation de la valeur professionnelle et l'instauration d'un régime indemnitaire en lien avec cette évaluation lui ont semblé contribuer à la modernisation de la gestion des ressources humaines des communes de Polynésie française. Nous conviendrons qu'il s'agit là de points positifs.

souhaité aller plus loin dans les objectifs de modernisation et d'attractivité de la fonction publique communale. Elle a ainsi modernisé la procédure de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés. Elle a également inscrit dans le statut général le recours au télétravail- vous évoquiez, monsieur le ministre, la spécificité du territoire polynésien, avec ses

Je souhaiterais attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'aider les communes à conserver- là encore, essentiellement pour des raisons de spécificités territoriales -les cadres qu'elles ont recrutés et formés. L'instauration du versement d'une indemnité par la collectivité d'accueil à la collectivité d'origine en cas de mutation d'un agent dans les trois ans suivant le recrutement pourrait, par exemple, constituer une réponse. Une telle disposition reviendrait du reste à s'aligner sur le droit commun de la fonction publique territoriale. C'est pourquoi nous avons du mal à comprendre le refus du Gouvernement d'accéder à notre requête. Par ailleurs, les modalités de réouverture du droit d'option permettant d'intégrer la fonction publique des communes de Polynésie française mériteraient d'être clarifiées. Dans un objectif de renforcement de l'attractivité de la fonction publique communale, il semblerait opportun d'étendre ce droit d'option, de façon explicite, aux agents contractuels ayant refusé la proposition d'intégration, ainsi qu'à ceux

de la rédaction actuelle. Enfin, pour renforcer les outils du dialogue social, la commission a étendu les compétences des comités techniques paritaires, par alignement sur le droit commun de la fonction publique. Ainsi, pour un certain nombre de sujets, la commission est allée plus loin que l'ordonnance initiale dans l'extension, à la fonction publique communale de Polynésie française, des dispositions en vigueur dans la fonction publique territoriale. Mes chers collègues, l'ordonnance du 8 décembre 2021, dans sa rédaction initiale, était quelque peu en deçà des attentes nourries depuis 2017. Nous avons donc souhaité l'enrichir et espérons qu'elle puisse contribuer efficacement à l'objectif ambitieux et nécessaire de modernisation du statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Polynésie française, ce sont 48 communes réparties sur 121 îles,

bien sûr prendre en compte les spécificités de tous les territoires, notamment de ses territoires ultramarins.

en 2017, il y a eu ce mouvement de grève par lequel les fonctionnaires et contractuels des communes de Polynésie française ont voulu exprimer leurs revendications.

et permettra quand la loi sera votée -de transposer un certain nombre de dispositions relatives à la fonction publique territoriale aux communes de Polynésie française. aussi, peut-être trop timidement dans certains domaines, d'adapter ces dispositions à un territoire dont j'ai dit succinctement- mais on pourrait être plus long -combien il avait de particularités. Ce texte comporte évidemment des aspects très positifs. Il renforce les prérogatives du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie et une commission consultative paritaires. Il favorise l'accès à la fonction publique communale.

Je pense aussi aux dispositions qui permettront de recueillir l'avis des commissions administratives paritaires en matière d'avancement et de mutation des personnels. Je pense encore aux pouvoirs accrus des comités techniques paritaires.

Aussi nous proposerons, par amendement, de rétablir les règles relatives à la déontologie et cette vigilance à l'égard des conflits d'intérêts.

était inscrit dans le texte initial que la valeur de la laïcité s'imposait au personnel des communes de Polynésie française,

permettant à tous de vivre ensemble, quelles que soient les convictions, les croyances ou l'absence de croyance des uns et des autres.

le 30 mai 2017, faisant suite au dépôt d'un préavis de grève dans l'ensemble des communes de Polynésie française, plusieurs réunions de concertation ont été organisées sur l'initiative du haut-commissaire de la République, avec les représentants de la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française, les élus représentant les communes au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et le président du Centre de gestion et de formation. Ces réunions ont abouti à un protocole d'accord, qui prévoyait, notamment, la mise en oeuvre d'un toilettage des textes de la fonction publique communale au regard des évolutions législatives intervenues en droit commun. Je profite de mon temps de parole pour saluer l'engagement constant et réel sur ce dossier de mon collègue Teva Rohfritsch, sénateur de Polynésie et rapporteur désigné sur le projet d'ordonnance lors de la consultation de l'Assemblée de la Polynésie Ce toilettage est nécessaire, au bénéfice des plus de 4 000 agents communaux de Polynésie, véritables chevilles ouvrières et garants du service public dans un territoire grand comme l'Europe, situé à plus de 15 000 kilomètres de Paris. En effet, le statut de la fonction publique des communes de la Polynésie apparaît, sur certains aspects, obsolète au regard des dernières évolutions législatives, notamment

ou plus récemment celle du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ainsi, par cette ordonnance de quarante-cinq articles, des avancées sont offertes aux agents dans les domaines de la mobilité, de la formation, des congés, de l'action sociale, de la mise à jour des procédures disciplinaires, du dialogue social, des obligations déontologiques, de la lutte contre les discriminations et, surtout, de la prévention des conflits d'intérêts.

Néanmoins, nous émettons de sérieuses réserves sur la suppression de la protection des lanceurs d'alerte en cas de dénonciation de conflits d'intérêts. La proximité entre les individus, censée fonder les différences de traitement des conflits d'intérêts, n'exonère en rien du respect de l'État de droit. La proximité entre les citoyens et les fonctionnaires doit se faire avec probité et un respect aigu des règles de transparence. De même, nous regrettons la suppression de la possibilité de recruter les fonctionnaires des communes sans concours, par la voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française. À ce titre, et sur ces deux sujets, nous voterons les amendements de rétablissement de la rédaction initiale de l'ordonnance proposés par le Gouvernement. Enfin, sur le contrôle déontologique, la proposition du Gouvernement donnant la possibilité à la commission de déontologie de saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et bénéficier de son expertise semble être le bon compromis entre l'application du droit commun et son adaptation aux spécificités locales. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte, nécessaire à la garantie, à l'efficacité et au bon fonctionnement des services publics polynésiens, que nous appelons de nos voeux et pour lequel nous oeuvrons sur l'ensemble du territoire français. Nous serons amenés à achever l'examen de ce texte d'ici à la prochaine législature. Dans l'intervalle, nous suivrons, aux côtés du ministre des outre-mer, les éventuels chantiers sur les sujets restant à traiter, en relation avec tous les acteurs concernés et dans l'intérêt total des Polynésiens.

étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette réforme du statut général des fonctionnaires communaux était attendue depuis longtemps,

et tient compte des évolutions législatives intervenues depuis 2011 dans le droit de la fonction publique territoriale. En outre, l'ordonnance du 8 décembre 2021 résulte d'une longue période de concertation entre le Gouvernement et les instances locales. C'est pourquoi je tiens à faire part de mon incompréhension et de ma déception quant au retrait soudain du projet de loi de l'ordre du jour, le 27 janvier dernier. En procédant ainsi, le Gouvernement balayait brutalement l'important travail mené depuis quatre ans.

L'objectif de l'ordonnance du 8 décembre 2021 est la valorisation des quelque 4 000 fonctionnaires communaux. Il s'agit de leur offrir un cadre juridique à la fois adapté et sécurisant. En premier lieu, l'ordonnance consolide les garanties dont disposent les fonctionnaires communaux en les alignant sur le droit commun de la fonction publique. En second lieu, elle conforte le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et apporte des assouplissements aux modalités de représentation des élus locaux

peut constituer un véritable handicap. Enfin, l'ordonnance modernise la gestion des ressources humaines des communes. À titre d'exemple, la notation est remplacée par une appréciation de la valeur professionnelle. De plus, les organes délibérants des communes et de leurs groupements ont la possibilité d'instituer un régime un régime indemnitaire lié à l'évaluation professionnelle. Si ce texte présente de nombreuses avancées, il ne reconnaît pas suffisamment les spécificités de la Polynésie française. cette prise en compte des réalités locales est indispensable. Je me réjouis donc des différentes initiatives prises en ce sens par notre collègue Lana Tetuanui. Je pense notamment à la suppression de l'inscription du principe de laïcité dans le statut général des fonctionnaires communaux. Le terme de neutralité semble effectivement plus approprié que celui de laïcité, d'autant plus que le droit applicable en Polynésie française a toujours appréhendé a toujours appréhendé la religion dans son contexte culturel particulier. C'est ainsi que la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'y a jamais été étendue. De même, eu égard aux réalités et particularités de la Polynésie, il n'est pas pertinent d'y créer un référent déontologue sur le modèle de la fonction publique métropolitaine. En effet, la probabilité que ce référent ait un lien personnel ou familial avec l'agent qu'il interroge est très forte. Pour toutes ces raisons, les élus du groupe Les Indépendants voteront ce projet

ont conduit à de grands mouvements sociaux en 2014 et surtout en 2017. Ce sont ces mouvements sociaux qui ont abouti à une concertation donnant lieu à l'ordonnance du 8 décembre 2021.

Oui, le Sénat peut s'honorer d'avoir maintenu à l'ordre du jour ce texte très attendu par nos compatriotes polynésiens. De la ratification des ordonnances, notre assemblée a débattu au début de ce mois

Ce gouvernement est celui qui a le plus utilisé les ordonnances. Pourtant, la part d'ordonnances ratifiées est, elle, en chute libre, tombant à 20 % pour l'ensemble du quinquennat.

Mais ne soyons pas dupes face à votre abandon coupable du principe constitutionnel de ratification expresse. Mes chers collègues, je reste particulièrement circonspect, pour ne pas dire ébahi ou abattu, face à la position du Gouvernement devant ce manque criant : il affirme « chercher à identifier, parmi les lois d'habilitation, les ordonnances qui nécessiteraient un débat, selon les voies et moyens que décideraient le Sénat et l'Assemblée nationale

Je tiens à saluer notre collègue Lana Tetuanui pour son engagement auprès de son territoire et pour les concertations qu'elle n'a cessé de mener sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui.

de votre jeu politique. L'urgence du terrain devrait vous obliger ; le travail des acteurs de terrain devrait vous obliger ; la compréhension de l'équilibre de nos institutions devrait vous obliger ! Puisqu'il n'en est rien,

Le gouvernement actuel a nourri ce discours, avec ses objectifs initiaux de réduction des effectifs et sa loi de transformation de la fonction publique. Contractualisation, privatisation, précarisation et réduction du dialogue social ont été au programme. Alors que la crise liée à la covid a mis un frein au dénigrement des fonctionnaires, il est primordial de reconnaître leur valeur au quotidien et de défendre leur place au côté du privé, qui n'a pas vocation à empiéter sur le public. Qu'ils soient de métropole ou de nos outre-mer, les fonctionnaires se sont unis pour dénoncer non seulement ces attaques, mais aussi leurs conditions de travail, qu'il s'agisse du gel du point d'indice, du rétablissement de la journée de carence ou des suppressions de postes. À l'affaiblissement général de leur pouvoir d'achat, les fonctionnaires grévistes de Polynésie ont ajouté des revendications précises, comme l'instauration d'une indemnité de départ volontaire, le maintien des droits acquis avant l'intégration dans la fonction publique communale ou encore des majorations de congés annuels spécifiques. La fonction publique des quarante-huit communes de Polynésie française est récente : elle a été organisée en vertu de l'ordonnance de 2005, donnant un statut de droit public à ses agents. Ce nouveau statut uniforme leur permet de bénéficier de droits similaires à ceux des fonctionnaires publics territoriaux de métropole et leur confère les mêmes obligations. Cette importante transformation statutaire nécessite des adaptations et des actualisations, comme celles détaillées dans l'ordonnance de 2021, dont la ratification nous est proposée

Comme le prévoit l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les règles relatives à la fonction publique communale relèvent de la compétence des autorités de l'État. L'extension de dispositions du droit commun en Polynésie nous conduit d'ailleurs à réfléchir aux limites de l'adaptation locale. L'examen en commission des lois a permis de modifier certaines dispositions qui nous avaient alertés, comme le recul de la compétence des instances de dialogue social. Il a également permis d'ajouter des mesures demandées localement, comme l'inscription dans le statut du télétravail. Certes, nous pouvons entendre l'argument avancé pour retirer du texte les notions de conflit d'intérêts et de laïcité. Mais, avec tout le respect que nous portons à nos concitoyens polynésiens et aux spécificités locales, nous ne sommes pas favorables à ces retraits.

qu'à une réelle prise en compte des spécificités locales. D'ailleurs, certaines revendications des représentants syndicaux n'ont pas été retenues. Néanmoins, cette ordonnance résulte d'un travail abouti, mené avec les acteurs locaux

des dispositions retenues permettent de valoriser la fonction publique communale, et la patte de la commission des lois a permis de revenir sur des mesures insatisfaisantes. Tout en rappelant ses limites, tout en soulignant la nécessaire revalorisation générale du statut de la fonction publique et des droits des fonctionnaires, nous considérons que ce texte est utile. Il permettra en effet de premières avancées, qui devront être complétées par un travail continu entre les acteurs locaux

est un moment attendu tant par les élus communaux de notre collectivité que par l'ensemble des 4 600 agents concernés, c'est-à-dire ceux soumis à ce statut, de création récente. Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler brièvement que les communes de Polynésie sont, dans le paysage institutionnel, des collectivités relativement nouvelles. En effet, quarante-cinq des quarante-huit communes existantes ont été créées par une loi de 1971 et n'ont commencé à fonctionner que vers la fin des années 1970. Certes, ces collectivités se sont substituées aux districts ; mais ces dernières structures n'étaient pas dotées de la personnalité morale. morale. Destinées avant tout à exécuter les décisions du gouverneur et de l'administration de l'État, elles ne disposaient que de quelques agents d'exécution. Depuis lors, heureusement, les choses ont bien changé. L'institution communale, dotée de compétences effectives, oeuvre au bien-être de nos populations, tout particulièrement

En effet, dans la très grande majorité de nos îles, il n'y a pas d'autre administration que l'administration communale. La collectivité d'outre-mer est certes déconcentrée, mais elle ne peut être présente dans toutes les communes. Bref- on l'aura compris -, ici plus qu'ailleurs, la commune est un rouage essentiel pour nos concitoyens. Toutefois, jusqu'en 2005, le personnel communal était soumis à un statut de droit privé qui différait d'une commune à l'autre.

; mais il a fallu attendre encore six années pour qu'il soit effectif. En effet, les textes d'application de l'ordonnance ne sont intervenus que tardivement. C'est pourquoi il a fallu reprendre l'ensemble de ce statut, qui, sans avoir été appliqué, était déjà devenu obsolète. C'est à la suite d'un large mouvement de contestation de la part des agents, au cours de l'année 2017, que fut prise la décision de toiletter ce statut afin de le rendre plus attractif tout en le modernisant. Ainsi, le Gouvernement avait déjà consulté la Polynésie française sur un projet d'ordonnance au cours de l'année 2018. Il me paraît important de rappeler ici les nombreux échanges entre les différents partenaires et les autorités parisiennes, et surtout l'important travail rendu par les élus et les représentants du personnel. Or, à la fin de l'année 2020, nous constations que ce projet n'était toujours pas adopté. C'est pourquoi, en mai 2021, à la demande des membres du Conseil supérieur de la fonction publique communale, j'ai déposé une proposition de loi visant à adapter et à moderniser le statut de la fonction de la fonction publique communale polynésienne. Toutefois, ignorant cette proposition de loi, le Gouvernement nous a fait parvenir en juillet 2021 un nouveau projet d'ordonnance afin que les principes de la fonction publique territoriale métropolitaine

Mais le 27 janvier, contre toute attente, le Gouvernement faisait machine arrière et retirait de notre ordre du jour ce projet de loi de ratification sans que l'on sache pourquoi.

Dans l'ensemble, tel a bien été le cas de l'ordonnance du 8 décembre 2021, dont certaines avancées sont à saluer. il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de ses dispositions ne respectent pas nos spécificités : c'est pourquoi nous sommes convenus d'amender plusieurs articles de ce texte. Mes chers

articles. Mes autres amendements ont, hélas ! été écartés par la commission des finances : ils sont tombés sous le coup de l'article 40 de la Constitution, qu'il s'agisse du droit d'option à l'ensemble des agents n'ayant pas encore obtenu le statut de la fonction publique communale ; de la possibilité pour nos communes de mettre en place un dispositif de départ anticipé pour certains de leurs agents, lequel est déjà applicable dans le droit commun

: qu'il s'agisse de l'ordonnance du 8 décembre 2021 ou du texte de notre commission, je salue l'important travail visant à associer les instances locales. Il était tout à fait nécessaire de moderniser le régime juridique des plus de 4 500 agents municipaux française, notamment pour accroître l'attractivité de cette fonction publique communale. Le groupe du RDSE est donc satisfait de cette volonté de valorisation du statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française. Il ne saurait y avoir de sous-fonction publique dans l'État français. Il convient donc d'actualiser ce statut au regard des évolutions législatives intervenues plus généralement dans la fonction publique territoriale.

ou encore le renforcement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Cependant, cette réforme impose aussi de trouver un équilibre avec les spécificités de ces territoires. Puisque la différenciation territoriale a enfin fait son entrée dans le droit commun des collectivités, nous apprécierions d'autant mieux qu'elle soit mise en oeuvre pour un territoire régi par l'article 74 de la Constitution. Il était aussi impératif

de neutralité seule, introduite en guise de substitution, nous semblant insuffisante. Chers collègues, nous sommes favorables au droit à la différenciation de nos territoires ultramarins, mais nous sommes encore davantage attachés au respect des valeurs et des principes de la République, qui doivent s'appliquer d'une manière harmonisée sur tout le territoire national. Cette réserve faite, notre groupe votera dans sa majorité en faveur de ce projet de loi.

qui peuvent survenir à tout moment. Nous nous devons, en tant que législateurs, de faire en sorte que, partout sur le territoire de la République,

comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Cette avancée en matière de transparence de la vie publique permet de renforcer la prévention de ces conflits et le contrôle exercé sur les agents et responsables publics, qui peuvent se retrouver dans des situations où leurs intérêts personnels se mêlent à l'exercice de leurs fonctions.

Il est légitime de demander la prise en compte des spécificités de la Polynésie française lorsque le Gouvernement et le Parlement sont amenés à légiférer sur des politiques qui s'y appliquent. Cependant, en l'espèce, au regard de la définition qui pose les limites du conflit d'intérêts, nous ne considérons pas que la lutte contre ces situations puisse être exclue du statut des fonctionnaires publics communaux polynésiens. L'argument de la proximité pourrait en outre être avancé en métropole ou dans d'autres endroits où s'applique déjà la législation en la matière.

maintenu ? C'est avec grand plaisir, monsieur le ministre, qu'au bénéfice de la déontologie je retire mon amendement au profit de celui de Mme Éliane Assassi.

Monsieur le ministre, dans une petite commune de cinquante habitants où les élus sont frères et soeurs, où l'agent de police municipale est le neveu du maire,

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement concerne les prestations sociales que les collectivités peuvent mettre en place pour améliorer les conditions de vie de leurs agents et de leurs familles. Ces prestations, qui peuvent être individuelles ou collectives, peuvent tout aussi bien concerner la restauration, l'enfance, les loisirs ou le logement. La commission des lois a restreint le champ de l'action sociale des collectivités de Polynésie française en supprimant les prestations en matière de logement.

si notre assemblée décidait de supprimer le mot « laïcité » figurant dans le texte initial. En effet, ce mot nous est cher.

l'idée de cet amendement n'est pas de revenir sur les particularités locales du territoire polynésien ni sur la non-application de la loi du 9 décembre

nettement supérieur à tous les autres principes.

intentions des auteurs de ces amendements identiques. En tant que législateur-

ces équilibres existent d'ores et déjà dans les territoires. Ils ont été construits depuis des centaines d'années, même des millénaires.

les principes, les us et les coutumes qui existent dans nos territoires. J'en appelle à la conscience de mes collègues sénateurs.

La création d'un référent déontologue dans les administrations publiques va dans le bon sens et offre aussi un nouveau droit aux fonctionnaires, celui de consulter une personne formée lorsqu'ils le souhaitent. En cas de doute, afin d'éviter de se retrouver dans une situation incompatible avec ses fonctions, le fonctionnaire dispose de ce nouveau moyen pour obtenir des conseils. L'ordonnance prévoyait d'étendre cette disposition aux membres de la fonction publique communale, mais la commission a voté un amendement supprimant cette extension,

moderniser ces modalités de recrutement en les alignant sur le droit de la fonction publique territoriale ; nous proposons, de plus, l'aménagement des modalités de déroulement des concours et des examens pour les candidats reconnus travailleurs handicapés. Dans un second temps, il conviendrait que cette disposition soit complétée, comme en droit commun, par la possibilité, pour les communes, de recruter des personnes handicapées en qualité d'agent contractuel, avant leur titularisation. nous avons donc du mal à comprendre pourquoi le Gouvernement s'oppose ainsi à un alignement sur le droit commun, lequel permettrait pourtant plus efficacement aux personnes handicapées d'accéder à la fonction publique communale, tout en offrant davantage de souplesse aux employeurs communaux. L'avis est donc défavorable. La parole est à

la création de cette nouvelle catégorie de congé avec traitement constitue une charge financière pour les communes ; d'autre part, les conditions dans lesquelles l'agent peut s'absenter pour participer à une activité de nature militaire ou en lien avec la réserve sont, selon nous, insuffisamment encadrées dans cet amendement. Par conséquent,

: c'est ainsi qu'il faut comprendre la laïcité dans la République ; c'est le vivre-ensemble qui vaut partout, dans tous les territoires de la République. Aussi est-ce avec plaisir que notre groupe votera ce texte.

texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.